sa position sur les garanties de l'État pour la construction d'établissements scolaires français à l'étranger. Or le Président de la République a annoncé son souhait de voir doubler le nombre d'élèves dans les établissements homologués

notamment lorsque l'État doit recapitaliser certaines entreprises- tel fut le cas d'Areva et de Dexia, il n'y a pas si longtemps. Dans la plupart des cas, les pertes financières sont absorbées par l'APE, il arrive qu'il faille les colmater en gestion, en faisant appel au budget général de l'État. C'est arrivé neuf fois entre 2009 et 2018, pour un montant cumulé de presque 34 milliards d'euros

financières de l'État qui auraient pour effet de faire perdre à l'État la majorité des titres ou les droits de vote d'une société. Il s'agit là d'une simple question de transparence. En outre, nous souhaitons que le Gouvernement informe le Parlement s'il a signé un pacte d'actionnaires

la Cour des comptes a recommandé de faire évoluer le statut de l'APE afin que celle-ci soit transformée en opérateur public doté de la personnalité morale, à charge pour cette dernière de verser chaque année un dividende au budget général de l'État correspondant à une part des produits des cessions réalisées et des dividendes qu'elle aurait elle-même perçus. Un premier rapport a été remis par le Gouvernement au Parlement sur ce sujet en 2018. Il s'agirait de le mettre à jour avec les données disponibles depuis 2018, dans un contexte de fortes privatisations et d'une affectation incertaine des recettes qui en sont tirées pour alimenter notamment le fonds pour l'innovation et l'industrie.

ainsi que par nos collègues à l'été 2018, en application de l'article 178 de la loi de finances pour 2018. Nous demeurons convaincus que le statut actuel de l'Agence des participations de l'État ne convient pas,

: La parole est à M. Jean-Yves Leconte. Le projet de loi de finances pour 2020 ne prévoit plus aucune autorisation d'avance pour l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), bloquant tout projet immobilier d'établissement en gestion directe, dont le financement n'est pas possible sur fonds propres.

en gestion directe. Il s'agit d'ouvrir une autorisation d'avances de 20 millions d'euros au profit de l'AEFE, afin qu'elle puisse financer des investissements immobiliers dans les établissements français à l'étranger.

». Vous entendez, cher collègue, renforcer les crédits alloués aux avances à des organismes distincts de l'État- ici à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, afin de l'aider à financer des projets. Or celle-ci a déjà bénéficié de six avances entre 2012 et 2018 et il lui reste à rembourser deux tiers des montants. la subvention pour charge de service public octroyée à l'AEFE au titre de la mission « Action extérieure de l'État » connaît une augmentation de près de 25 millions d'euros.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, mon intervention portera exclusivement sur les crédits de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines Dotée de 10,5 milliards d'euros en 2020, cette mission porte les crédits des deux grandes administrations de Bercy, que sont la direction générale des finances publiques (DGFiP) et la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI),

hausse des dépenses publiques. Vous tous ici savez que ces deux administrations de réseau sont essentielles pour nos territoires. Elles sont pourtant confrontées à de nombreux défis. J'en citerai trois.

Le Gouvernement avait appelé à un changement de méthode ... Il a envoyé à chaque élu local, chaque député et chaque sénateur, une carte des futures implantations de la DGFiP dans son département. Curieuse manière d'entamer une négociation ! Nous espérons néanmoins que ces négociations aboutiront à un consensus local.

dernières n'ont que peu de temps pour candidater et le processus semble réservé aux villes moyennes. Comble de l'ironie, l'État exige que des surfaces immobilières soient mises à disposition de ses services au

dans les villes dynamiques et en pleine expansion. Nous rencontrons la même problématique pour les maisons France services. Qui peut nous garantir que les collectivités territoriales ne seront pas mises à contribution pour des services que l'État doit lui-même assurer ? Monsieur le secrétaire d'État, sans doute pourrez-vous nous apporter des précisions sur ce point.

et que ces administrations sont écrasées par leur dette technologique au point qu'elles doivent recourir à la mission « Action et transformation publiques » pour financer leurs projets innovants. Cette dette technologique est insoutenable et provoque son propre effet boule de neige : happés par la maintenance, ces crédits, mêmes supplémentaires, ne vont que très peu vers l'investissement et la création. Le troisième et dernier défi à relever par les administrations fiscale et des douanes est la transformation de leurs métiers, et leur capacité à faire face aux projets de restructuration.

Il faudra bien pourtant aborder cette question, ne serait-ce que pour donner davantage de visibilité aux agents des finances publiques et aux douaniers. il me revient de vous exposer la position de la commission des finances, qui a adopté les crédits de la mission amendés. Elle y est donc favorable. Ce faisant, elle manifeste son soutien aux efforts de rationalisation et de modernisation de ces administrations.

Nous espérions des progrès ; cela ne semble pas être le cas. Je suis surpris de constater qu'une mission qui est supposée aller vite et participer à la transformation de nos administrations mette autant de temps avant d'atteindre sa pleine vitesse d'exécution. Claude Nougein et moi-même avons pu noter que les fonds prévus dans les différents programmes de la mission venaient, dans les faits, compenser l'insuffisance des crédits inscrits sur les programmes traditionnels. Cela explique que le critère de sélection des projets, fondé sur les économies attendues, ait été partiellement abandonné. la commission des finances souhaite s'en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée. Il nous semble, en effet, qu'elle relève davantage d'un affichage politique, d'une stratégie de communication que d'un réel effort budgétaire.

pour une valeur comptable estimée à 63 milliards d'euros. Il est pourtant mal géré et victime de la faiblesse de la direction immobilière de l'État (DIE) à l'échelon interministériel. Je rappelle que la DIE est sans pilote depuis l'été dernier. Ce CAS a vocation à financer les opérations structurantes et d'entretien lourd du patrimoine immobilier de l'État.

résulte un déficit répété et un défaut d'entretien, malgré un rebond attendu en 2019. Pour toutes ces raisons, la commission des finances recommande depuis plusieurs années de diversifier les modes de valorisation du patrimoine immobilier de l'État.

éclairer. Nous considérons que les crédits consacrés par le CAS au Grand plan d'investissement relèvent de l'affichage. Les dépenses sont censées participer à la transition énergétique par la rénovation des bâtiments, mais nous n'avons aucun indicateur en Pire encore, l'administration n'est pas capable de définir avec précision le montant des crédits consacrés à ces travaux de performance énergétique ! Vous admettrez, monsieur le secrétaire d'État, que nous sommes encore loin du « budget vert

à hauteur de 16 millions d'euros pour 2020. Il est satisfaisant de constater que les crédits correspondant à la revalorisation du barème de remboursement des frais de repas aient été répartis en seconde délibération à l'Assemblée nationale. En revanche, vous en conviendrez, monsieur le secrétaire d'État, il était surprenant que ces crédits fussent inscrits au au titre 2 alors qu'ils concernaient des dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel. Quand aura lieu la répartition des crédits relatifs à la revalorisation du régime indemnitaire des agents de la filière sociale, prévus pour 2020, ainsi que celle des 24,7 millions d'euros restés inscrits pour l'année 2019 ?

dont le déséquilibre démographique rend la contribution solidaire de l'État obligatoire. Il s'agit principalement de ceux de la SNCF et de la RATP, qui absorbent les deux tiers de la contribution, mais aussi de ceux des mines et des marins.

Un régime est dit « fermé », lorsqu'il n'accepte plus de nouveaux cotisants. C'est le cas de la Seita, de l'ORTF et de la SNCF dès cette année, en raison de l'entrée en vigueur de la réforme ferroviaire. Pour 2020, la contribution de l'État sera de 6,2 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes spéciaux déficitaires, en baisse de 56 millions d'euros, ce qui correspond à la sortie du régime de retraite complémentaire des exploitants agricoles. Globalement, la contribution est stable, car les régimes fermés dégagent des économies qui compensent les hausses de subvention à la RATP et du congé de fin d'activité des transports routiers. Nous nous inquiétons de l'impact du Brexit sur le régime des marins, qui n'est pas provisionné et qui pourrait pourtant être colossal. Dans un contexte de réforme, il m'importe particulièrement de relever que les subventions de l'État censées compenser le déséquilibre démographique financent aussi des avantages spécifiques. La Cour des comptes a estimé qu'il s'agit de 400 millions d'euros annuels pour la RATP

Pour mémoire, entre 2010 et 2018, le niveau des pensions a augmenté de 16 % à la RATP, de 12,5 % à la SNCF, mais de seulement 1,8 % dans la fonction publique territoriale On peut légitimement se demander pourquoi la solidarité nationale finance des avantages aussi spécifiques que substantiels. Si chaque régime spécial a un fondement légitime et une histoire, il est de notre responsabilité de subvenir à leurs besoins, mais aussi d'en fixer les limites, eu égard au respect de l'utilisation des fonds publics. Très bien ! Le compte d'affectation spéciale « Pensions » retrace les opérations relatives aux pensions civiles et militaires de retraite et d'invalidité des agents de l'État 59,6 milliards d'euros sont prévus pour 2020, les dépenses progressant, comme les recettes, de 1 %. La revalorisation des pensions sera différenciée, soit 1 % pour les pensions inférieures à 2 000 euros et 0,3 % pour celles qui sont supérieures à cette somme. Les recettes du CAS progressent moins que la masse salariale de l'État en raison des primes généralement non cotisées, mais aussi du fait de la déformation de l'emploi public. Depuis 2008 le nombre de contractuels a considérablement augmenté, tandis que le nombre de cotisants au régime de la fonction publique d'État a diminué de 11,8 %. Dans ce contexte salarial, la nouvelle augmentation du taux des cotisations salariales n'apporte pas beaucoup de nouvelles recettes, mais les cotisations supportées par les fonctionnaires sont aujourd'hui quasiment équivalentes à celles des salariés du régime général. Quant à la part des primes dans l'emploi public, elle est de 42,3 % pour les cadres A+, 33,9 % pour les policiers et 12,6 % pour les enseignants. J'appelle votre attention sur cette disparité et l'évidente complexité à faire converger des droits, si, demain, dans le cadre de la réforme, les primes entrent dans la base de cotisation des retraites. Il faudrait alors convertir les droits actuellement constitués dans les droits du nouveau régime. Pour les fonctionnaires, c'est techniquement impossible, puisque le service des retraites de l'État ne dispose pas des informations sur les primes versées dans le passé. présent en effet, ces primes n'entraient pas en compte dans le calcul de liquidation des droits. Au-delà des six derniers mois, on ne dispose donc pas de la mémoire des informations concernant la rémunération des fonctionnaires ! Je vous laisse imaginer les années de travail nécessaires pour reconstituer les carrières. Nous avons donc là deux problèmes majeurs : l'obstacle technique pour recueillir les informations et le délai de transition nécessaire pour maintenir les droits attendus sans les décapitaliser ! Je termine en évoquant le solde général du CAS « Pensions le surplus de recettes sur les dépenses devrait dégager 1,4 milliard d'euros en 2020 et le solde cumulé serait alors de 9,4 milliards d'euros. Cet excédent pourrait atteindre 30 milliards d'euros en 2030, ce qui fait du CAS « Pensions » un contributeur majeur à l'équilibre du système de retraite global. Au terme de ces observations, compte tenu des nécessaires contributions de l'État aux régimes spéciaux et de la bonne tenue du CAS « Pensions », la commission des finances vous propose l'adoption des crédits de la mission. La parole est à M.

Ainsi, de 2013 à 2018, les sommes recouvrées par le contrôle fiscal ont baissé de 20 %, passant de 10 milliards d'euros à 7,8 milliards d'euros. Fraude à la TVA, aux cotisations sociales et, bien sûr, évasion fiscale sont au premier rang de ces comportements profondément antirépublicains.

Le budget qui nous est soumis poursuit ce triste effort en programmant 1 471 suppressions de postes entre 2019 et 2020. Ainsi, un tiers des emplois détruits dans la fonction publique d'État le seront dans l'administration de Bercy. Alors que le mouvement social des « gilets jaunes » a porté une exigence de justice fiscale, partagée par une très large majorité de l'opinion publique, vous baissez la garde, malgré vos propos enjôleurs, face aux principaux artisans de cette fraude fiscale massive : les plus riches et les grandes entreprises. Ce ne Ce ne sont certainement pas vos annonces en matière de contrôle aléatoire sur internet- contrôle par ailleurs susceptible de remettre en cause les libertés publiques -qui inverseront la tendance, pas plus que le transfert anarchique des moyens humains vers la sacro-sainte informatique.

également, à l'occasion de la sortie de ce rapport, que le Comité national de lutte contre la fraude ne se réunit plus et que le poste de Délégué national à la lutte contre la fraude est toujours vacant.

Mon département, la Seine-Saint-Denis, où il faudrait tout faire pour maintenir et développer les contacts humains, n'a pas été épargné, avec le regroupement des trésoreries de La Courneuve et d'Aubervilliers ou de Montreuil et de Bagnolet. Mon ami Jean-Paul Dufrègne signalait,

La dématérialisation- l'un des mots sacrés de votre start-up ! laisse de côté les plus fragiles. Miser sur le tout informatique est un facteur puissant de déshumanisation, et donc d'injustice et d'inégalités devant l'impôt, alors que le Défenseur des droits rappelait en janvier qu'il fallait respecter, en la matière, les principes fondateurs du service public : adaptabilité, continuité et égalité. Actuellement, 460 maisons de services au public, qui regroupent,

Cette hémorragie participe grandement à la désertification des territoires ruraux, mais aussi à la fragmentation sociale dans les quartiers populaires. Monsieur le secrétaire d'État, il faut mettre un terme à cette politique dictée par vos dogmes libéraux, pour accompagner

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui les crédits des missions « Gestion des finances publiques et des ressources humaines », « Action et transformation publiques » et « Régimes sociaux et de retraite ».

Une chose est devenue certaine : les Français ne font plus confiance à leurs régimes de retraite. Ils savent que les mutations démographiques de notre société obligent à une refonte en profondeur du système. Ils ont compris, et pour la plupart accepté-

Le Gouvernement a fait le choix courageux de réformer les régimes spéciaux, vache sacrée de toutes les organisations syndicales et de certaines organisations politiques, qui sonnent à nouveau le branle-bas de combat en criant à la casse sociale. C'est jouer sur les inquiétudes, du reste légitimes, de nos concitoyens, et ce alors même qu'aucun projet de loi n'a encore été présenté. On pourrait appeler cela une grève préventive. ! Les chiffres sont pourtant têtus et ne se laissent guère intimider par la mobilisation de jeudi, quelle que soit son ampleur. La mission « Régimes sociaux et de retraite », qui regroupe les subventions d'équilibre versées par l'État à dix régimes spéciaux de retraite, notamment ceux de la RATP et de la SNCF, sera dotée de plus de 6 milliards d'euros en 2020. Les crédits programmés pour équilibrer ces régimes augmentent encore cette année. On est donc loin de la casse sociale dont on nous rebat les oreilles. de la gestion des ressources humaines de l'État : les crédits de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines », qui concernent essentiellement l'administration fiscale et l'administration des douanes, se stabilisent entre 2019 et 2020, 2020, bien loin des coupes sèches dans les effectifs des services publics qui sont évoquées çà et là. Certes, la diminution des effectifs de la mission se concrétise par la baisse du plafond d'emplois de quelque 1 500 équivalents temps plein travaillé entre 2019 et 2020. C'est la DGFiP qui contribue principalement à cet effort ; il est bon que Bercy prenne les devants et montre l'exemple pour diminuer les effectifs dans la fonction publique, même si les baisses de dépenses de personnel ne représentent guère qu'un demi-point en volume. Cependant, nous sommes nombreux dans cette assemblée à regretter que le Gouvernement ait renoncé à ses objectifs de réduction des effectifs dans la fonction publique, singulièrement dans la fonction publique d'État.

C'est trop peu ! La contraction de la fonction publique aura donc essentiellement été supportée par les collectivités territoriales. Il est facile de pointer du doigt ce rétropédalage : le Gouvernement en a pris le risque en se fixant des objectifs chiffrés. la focalisation sur de tels objectifs ne doit pas nous faire perdre de vue l'essentiel : personne ne désire réduire des effectifs pour réduire des effectifs, mais tout le monde devrait souhaiter que notre fonction publique devienne chaque année plus efficiente. C'est pourquoi nous entretenons encore les espoirs que nous avions placés dans la mission « Action et transformation publiques », créée en 2018. Nous portons ainsi un regard bienveillant, quoique vigilant, sur l'augmentation de près de 40 % des crédits qui lui sont alloués. Nous regrettons, toutefois, que les ambitions d'économies affichées par le Gouvernement dans le cadre du projet Action publique 2022 soient revues à la baisse. Nous espérons que ces crédits contribueront tout de même à transformer l'administration et à renouveler le service public, notamment selon les deux priorités que sont la transition énergétique et la transition numérique de l'État. la transition numérique de l'État. Le mouvement engagé par le Gouvernement se heurte donc à la réalité et subit la résistance de l'État, qui semble toujours se soustraire à toute bonne volonté de rationalisation. Le principe de réalité commande de revoir à la baisse l'allure de la réforme, comme un marcheur à qui l'on annoncerait qu'il devra parcourir la même distance, dans le même temps, mais en avançant les deux pieds dans l'eau. Pour ces raisons, le groupe Les Indépendants salue la démarche entreprise par le Gouvernement, mais regrette, vous l'aurez compris, que son rythme ne soit pas plus rapide. La parole est à M. Jean-Claude Requier.

et l'administration fiscale correspond, à elle seule, à 80 % des effectifs. Dès lors, ne pourrait-on pas envisager un intitulé plus explicite ? Les défis

En parallèle, l'État regroupe les différents services publics, tous ministères confondus, au sein des maisons de services au public, qui représentent un enjeu considérable d'accès au service public dans de nombreux territoires. pratique, toutefois, les fermetures de trésoreries- les perceptions, comme on dit chez nous -ne vont pas sans susciter des inquiétudes de la part des particuliers comme des agents de ces structures. Pour se faire une idée fidèle de la réorganisation, il faut étudier la situation dans chaque territoire.

subisse coup sur coup plusieurs fermetures de services publics. C'était là, je le rappelle, l'un des enjeux de la création de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, que nous avons portée ici même

d'un point de vue budgétaire, la mission comprend le programme « Fonction publique », qui vise le budget de l'ENA et des instituts régionaux d'administration, pour un ensemble d'environ 80 millions d'euros. À ce sujet, nous attendons, avec une impatience non feinte, les conclusions de Frédéric Thiriez, du rapport a été reportée au mois de janvier. Par ailleurs, l'analyse des crédits de la mission « Régimes sociaux et de retraite » et du compte d'affectation spéciale relatif aux pensions des fonctionnaires montre que, si les retraites des régimes spéciaux restent encore subventionnées dans des proportions importantes, leurs situations, au demeurant très diverses, tendent à converger vers le régime général. Il faut le relever, car le maintien de ces régimes sera au coeur

sur l'absence de politique immobilière unifiée, sur les conséquences de la cession de certains actifs, sur le coût de la location de locaux, avec une hausse de plus de 6 % des loyers en 2018, sur les biens restants, plus difficiles à céder, etc. La contribution du parc de l'État à la transition énergétique pourrait, et devrait, constituer un axe stratégique majeur. En conclusion, monsieur le secrétaire d'État, le groupe du RDSE votera évidemment les crédits de ces quatre missions et de ces deux comptes d'affectation spéciale, dont les enjeux ne sont peut-être pas les plus médiatiques, mais qui contribuent, à n'en pas douter, à moderniser l'État et nos services publics, au plus près des besoins et des attentes de nos concitoyens.

par l'adoption de la loi de transformation de la fonction publique. L'objectif de cette loi était de moderniser le statut et de renouveler les conditions de travail en simplifiant l'architecture des instances de dialogue et en rassemblant un certain nombre de missions. Elle a assoupli les modalités de recrutement des agents publics en ouvrant davantage de postes aux contractuels et elle a mis en place le CDD de projet, qui permet la mobilisation de compétences externes pour la conduite et la mise en oeuvre d'un projet. Les collectivités pourront ainsi bénéficier de personnels à haut niveau de compétences pour mener un chantier d'équipement, de développement ou d'urbanisme à caractère exceptionnel. Cette simplification s'est accompagnée de garanties création d'une prime de précarité applicable aux contrats de courte durée, renforcement des parcours de formation, exonération du jour de carence pour les femmes enceintes, renforcement de l'accompagnement individualisé des fonctionnaires reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

de la conformité avec la réglementation en vigueur. Sur cette base, le ministre du budget et des comptes publics a annoncé en mars dernier la mise en place d'un cadre rénové entre les entreprises et l'administration baptisé « nouvelle relation de confiance ». Parmi les mesures prévues figurent l'accompagnement fiscal personnalisé pour les PME, l'identification des sujets fiscaux dont le traitement mérite d'être clarifié, les options fiscales qui s'offrent à l'entreprise, le tout pouvant donner lieu à un rescrit opposable à l'administration fiscale. L'action de l'administration se tourne ainsi davantage vers le conseil et moins vers la sanction. Il faut adapter le service public aux transformations économiques, au numérique, à l'intelligence artificielle, ainsi qu'aux attentes des usagers, comme l'ont fait les entreprises. C'est donc la fin d'un modèle standardisé et uniforme. Le service public doit être plus personnalisé et plus ouvert et, à cette fin, renoncer à une forme de gestion centralisée, uniforme et descendante.

: nous n'avons pas la même conception de la gestion ! Lors de la présentation du plan Action publique 2022, le Premier ministre souhaitait réformer la fonction publique selon trois objectifs : alléger, simplifier, rapprocher du terrain. Il a mille fois raison.

fiscaux, la mise à jour automatique des situations fiscales- un pas vers la simplification de l'impôt, à laquelle le groupe Union Centriste est particulièrement attaché -, la création d'un guichet unique national de dédouanement, qui va aussi dans le sens de la dématérialisation et, enfin, la création de maisons France services dans chaque canton d'ici à 2022, qui représente un progrès considérable. Mon groupe ne peut que se réjouir de cette initiative, qui favorise un rapprochement entre les services et les usagers. Il ne faut jamais oublier que, si l'État peut gouverner de loin, il ne peut le faire correctement que de près. Néanmoins, si ces avancées sont louables, notamment en matière de modernisation de la fonction publique, il reste à opérer l'essentiel : le travail relatif au nombre de fonctionnaires.

la valeur comptable de l'ensemble du patrimoine immobilier de l'État dépasserait 63 milliards d'euros,

qui concerne la SNCF, systématiquement montrée du doigt comme expression de la pseudo-aberration de notre système, son régime spécial connaîtra dès l'année prochaine une évolution décisive, à la suite de la réforme mettant fin au statut des cheminots. Dramatiser cette problématique et plaider l'extinction plus rapide du régime sont un véritable piège.

De plus, les réformes successives ont contribué à la banalisation de ces régimes spéciaux, pour les adapter aux nécessités de la société contemporaine. Ainsi, je rappelle que la dernière réforme des retraites, celle de Marisol Touraine, touche aussi ces régimes spéciaux, puisque le nombre d'annuités est passé à quarante-trois pour tout le monde pour la génération 1973. De fait, cette réforme joue sur l'augmentation de la durée de cotisation pour tous les salariés, quel que soit leur régime : désormais, pour les générations nées à partir de 1958, ce paramètre augmentera d'un trimestre tous les trois ans à partir de 2020, pour atteindre quarante-trois Par ailleurs, les travailleurs entrant dans la vie active et encore susceptibles de bénéficier de ces régimes spéciaux ne dérogent pas à la règle commune. Ils entrent eux aussi plus tard dans la vie active : le bénéfice qu'ils tirent du système actuel s'éteindra donc rapidement. ce sont les caractéristiques propres de ces régimes qui intéressent le Gouvernement, à des fins d'instrumentalisation. Pourtant, chacun d'entre eux est le fruit de luttes et de négociations liées à des conditions de travail particulières. Ils font partie d'un édifice social que certains se plaisent à décrire comme baroque, mais qui trouve son sens au regard de l'histoire et des conditions de travail de leurs bénéficiaires. En tout état de cause, de cause, passer à un système à points n'éteindrait pas du jour au lendemain les régimes spéciaux concernés, et l'État devrait continuer à débourser des sommes importantes pendant un certain temps. Dans son entreprise radicale de réforme, l'exécutif a sollicité le Conseil d'orientation des retraites le Premier ministre lui a demandé de lui fournir un état de la situation financière de l'actuel système de retraite à l'horizon de 2030 et d'éclairer les voies et moyens d'un équilibrage financier en 2025. L'espoir du Gouvernement était de voir établir que des mesures de correction s'imposeraient avant 2025, date envisagée pour la mise en oeuvre de la retraite par points. Or, dans l'introduction de son étude, le précise bien : « Le fait que ce rapport présente l'impact chiffré de potentielles mesures ne signifie pas que celles-ci soient considérées comme opportunes par tous. » Alors que la nouvelle concertation devait s'appuyer sur son rapport, cet organisme a fait l'objet d'une attaque en règle par le président de l'Assemblée nationale,

qui, elles-mêmes, déclinent différents scenarii. En d'autres termes, quelle que soit sa rigueur, extrême, cet organisme ne peut pas prédire l'avenir ; la finesse de ses projections et leur diversité ne peuvent être assimilées à une capacité de divination. On lui demande de soumettre des hypothèses, c'est ce qu'il fait.

On peut donc se poser la question du remplacement d'un système complexe, mais qui fonctionne, par un autre, en apparence plus simple, mais dont les effets demeurent largement méconnus. Ce propos ne procède pas d'une volonté de ne jamais rien changer : nous demeurons mobilisés pour la mise en place du système le moins producteur d'inégalités possible. Mais nous ne sommes pas prêts à donner un blanc-seing au Gouvernement sur un projet qui plonge la société française dans un climat anxiogène dont elle n'a pas besoin

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je vous prie d'excuser mon retard. Le projet de loi de finances pour 2020 semble enregistrer l'abandon de l'objectif de suppression de 50 000 équivalents temps plein dans la fonction publique d'État, comme le Président de la République l'a laissé entendre au sortir du grand débat. Vous-même, monsieur le secrétaire

L'avis budgétaire « Fonction publique » porte prioritairement sur la fonction publique d'État, plus précisément sur le programme 148, destiné à compléter les actions des ministères en matière de ressources humaines. Ce programme est doté de 211,21 millions d'euros, un montant en hausse de 2,74 % par rapport à 2019.

qui poursuit la mise en oeuvre de son plan de transformation pour revenir à l'équilibre budgétaire en 2020 et dont la subvention s'établit à près de 30 millions d'euros. Le budget de l'action sociale interministérielle s'établit à 126 millions d'euros, en hausse de 6,23 %. Trois aides concentrent plus de 80 % des crédits : les chèques vacances, les chèques emploi service universels et les places en crèche. Il est regrettable que, depuis 2019, les aides pour le recrutement d'apprentis dans la fonction publique d'État ne figurent plus dans le programme 148, mais soient réparties dans les budgets des différents ministères, ce qui amoindrit leur lisibilité. Néanmoins, la commission des lois a émis un avis favorable sur les crédits du programme 148. Plus largement, je souhaite évoquer l'organisation des concours administratifs, qui, conformément au statut, demeurent la voie d'accès traditionnelle à la fonction publique, malgré la loi de transformation de la fonction publique.

sur une plateforme les coordonnées et les profils des membres de jury, en prévoyant des épreuves mutualisées entre plusieurs concours pour faciliter la conception et la correction des sujets et en généralisant généralisant la dématérialisation des corrections. Par ailleurs, comme aux concours des IRA et de l'ENA, des épreuves pratiques et des épreuves collectives de mise en situation pourraient être proposées. Le calendrier des concours pourrait être publié sur le site « Place de l'emploi public », qui regroupe déjà les offres d'emplois

À la suite de sa mise en oeuvre réussie, le prélèvement à la source poursuit son déploiement, parallèlement à d'autres projets de transformations majeurs tels que la suppression définitive de la taxe d'habitation, la fin du paiement en numéraire et la déclaration tacite.

Nous allons aussi mettre à profit 2020 pour mener des travaux de modernisation de la gestion budgétaire et comptable, renforcer la performance des chaînes d'achats et de dépenses. L'expérimentation d'unification de la chaîne de la dépense, engagée cette

Ces réformes sont conduites en prenant en compte plusieurs priorités. Notre objectif premier sera de renforcer la présence et l'accessibilité des services publics sur le territoire. Nous avons proposé une réforme de l'organisation territoriale de la DGFiP, avec la volonté d'augmenter de 30 % le nombre de lieux d'accueil offerts par cette direction.

Nous souhaitons aboutir à des cartes cibles et des conventions pluriannuelles, pour que la présence de l'État dans les territoires à travers la DGFiP soit stabilisée et qu'une lisibilité soit offerte aux élus, aux agents, aux organisations syndicales et aux territoires. Nous nous appuierons évidemment sur le réseau des maisons France services

Nous devons prêter une attention particulière à la question de l'accès aux services numériques, en ayant à l'esprit que 13 millions de nos concitoyens en sont éloignés, faute soit de réseau soit de pratique. D'où l'importance d'une présence humaine et du maintien d'une médiation pour garantir l'accès aux services.

été en 2018, 350 en 2019 et 100 le seront en 2020. Hors crédits de personnel, 20 millions d'euros ont été alloués sur la période 2018-2022 pour l'équipement des nouveaux agents et les évolutions informatiques et immobilières rendues indispensables par le rétablissement de la frontière. En ce qui concerne le fonctionnement interne du ministère, nous souhaitons préserver nos capacités à accompagner la transformation et à moderniser nos outils de travail. De ce point de vue, nous partageons la nécessité, soulignée par les deux rapporteurs spéciaux, MM. Nougein et Carcenac, d'être attentif aux attentes du personnel. C'est le sens de la consultation que nous avons lancée auprès des agents pour élaborer une feuille de route en matière de simplification et d'amélioration des conditions de vie au travail, donc aussi de l'efficacité des services. Entre autres outils destinés à améliorer la qualité de vie au travail,

et de la fonction publique est en cours, et nous respecterons les dates arrêtées par le Parlement, puisque l'ensemble des mesures applicables en 2020 feront l'objet de décrets d'application au plus tard

complémentaire, le Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État finance le développement de produits et services numériques innovants. Nous continuerons de le mobiliser en 2020, pour réussir le passage à l'échelle de cette dynamique nouvelle.

se moderniser, leur restructuration, leur réorganisation et la mobilité de leurs agents. Nous veillerons à ce que la future agence de reconversion et de reclassement puisse le mobiliser plus aisément.

d'être indiqué, cet amendement vise à geler, pour les six premiers mois de l'année, l'évolution des dépenses relatives au GVT et les mesures de revalorisation. Il est vrai que la maîtrise de la masse salariale de l'État constitue un enjeu fondamental pour l'assainissement de nos finances publiques.

dispose que les fonds des personnes hébergées dans un établissement public de santé, social et médical-social et faisant l'objet d'une mesure de protection juridique du fait de leur état de santé ne leur permettant pas d'assumer les actes de la vie quotidienne seraient dorénavant,

Quel est l'avis de la commission ?

pour revenir vers l'équilibre. Cela explique aussi les variations d'une année sur l'autre des crédits accordés par l'État.

Ce régime, héritage des luttes sociales, est la contrepartie imparfaite du sacrifice des hommes et des femmes qui ont oeuvré à la prospérité nationale. Certes, depuis un décret de 2011, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ne compte plus de nouveaux affiliés, et ses ressortissants s'éteignent progressivement, avec une moyenne d'âge particulièrement particulièrement élevée, au-delà de 80 ans. Depuis plusieurs années, la baisse des crédits alloués au régime des mines, en particulier à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), et son volet action sanitaire et sociale est constante. Mais la diminution annuelle de 5 % du budget ne tient pas compte des besoins de cette population, justement vieillissante. Entre 2017 et 2018, ce sont même 10 % de baisse des dotations qui ont été enregistrés, sans aucune corrélation avec une évaluation des besoins grandissants de la population concernée. En conséquence, En conséquence, l'ANGDM, en tant qu'opérateur actuel chargé de gérer l'action sociale, s'est vue dans l'obligation de stopper certains versements ou prestations dans un contexte de tensions en interne, tandis que les manques cumulés de budget des années précédentes obèrent déjà les comptes 2020. Nous proposons donc par le biais de cet amendement de corriger cette baisse des moyens, afin de garantir la compensation des besoins et d'assurer les rattrapages, estimés par les syndicalistes. Cette mesure vise à rétablir une justice envers les anciens mineurs et, surtout, envers leurs veuves, qui sont déjà lourdement affectées par la fin de la demi-part fiscale, l'augmentation de la CSG et par un niveau de pension particulièrement faible. Pour l'ensemble de ces raisons, à travers cet amendement, il s'agit d'envoyer un signal volontaire,

? Cette décristallisation intervient bien tardivement. Il serait intéressant de savoir combien l'État a pu économiser jusqu'à présent. L'avis de la commission des finances serait favorable sans réserve si la posait pas une difficulté juridique- mais sans doute le Gouvernement va-t-il la lever. En effet, je ne suis pas certaine que les dispositions relatives à la CNRACL, qui devra prendre à sa charge le supplément des pensions, ainsi que le précise l'exposé des motifs de l'amendement, relèvent pleinement du domaine des lois de finances. J'émets donc un avis de sagesse